Il s'agit de prendre en compte, dans le calcul de la valeur locative moyenne, le fait que les établissements d'enseignement scolaire pratiquent assez fréquemment le commodat ou la location à l'euro symbolique. Or la direction

ce qui existait depuis très longtemps, à savoir la pratique du commodat dans l'enseignement sous contrat. Cela concerne naturellement toutes les confessions. Je rappelle que, dans un certain nombre de secteurs, ces établissements remplissent une véritable mission de service public, soit parce qu'ils offrent des formations qui ne sont pas disponibles dans l'enseignement public,

les échanges se poursuivent pour que,, soit ajustée la prise en compte des valeurs foncières des différents locaux en fonction de la répartition de leur usage. Il ne me semble donc pas utile à ce stade de fixer dans la loi les dispositions que vous proposez. La parole est à Mme Christine Lavarde,

à jour s'effectue à partir de l'évolution annuelle des loyers commerciaux sur la base des tarifs 2017 non revalorisés. La perte pour l'ensemble des collectivités se monte à 140 millions d'euros. Cet amendement vise à rectifier ce

Lorsque la décision a été prise de reporter l'application de la révision d'un an, de 2018 à 2019, il a été décidé dans le même temps d'appliquer un coefficient uniforme de revalorisation à caractère exceptionnel pour éviter que le report ne se traduise par une année blanche en termes de dynamisme des bases.

Cette prorogation entend poursuivre et maintenir l'effort de soutien au secteur de la presse. En second lieu, la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a apporté plusieurs ajustements à ce dispositif exceptionnel, créé par la loi du 17 avril 2015 portant diverses le bénéfice de cette réduction d'impôt temporaire a notamment été élargi aux versements afférents aux souscriptions au capital de sociétés d'amis ou de lecteurs regroupant exclusivement des actionnaires individuels et dont l'objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d'une entreprise de presse. Toutefois, le texte ne permet pas une bonne application de cet élargissement à l'investissement indirect, dans la mesure où la loi n'exige pas explicitement que les sommes versées à ces sociétés soient effectivement employées dans des entreprises de presse, contrairement à ce qui est Dès lors que l'avantage fiscal ne se justifie que s'il permet de mobiliser effectivement des sommes pour renforcer les fonds propres des entreprises de presse, le présent amendement vise à conditionner le bénéfice de cet avantage fiscal à l'affectation effective des versements

Cet avantage fiscal nouveau vise à inciter au financement privé des structures spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l'écoute et l'orientation des victimes de violences sexuelles et sexistes. Cet amendement répond en partie à l'appel formulé par la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, pionnière en la matière, en faveur de la multiplication de telles structures. Le développement de ce modèle a de permettre la couverture de l'ensemble du territoire par un accueil adapté à la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences sexuelles durant l'enfance, à l'instar des mutilations génitales féminines, ou durant l'âge adulte. adulte. La Maison des femmes de Seine-Saint-Denis fonctionne essentiellement grâce aux dons des personnes privées. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose une incitation fiscale spécifique. Il s'inspire également des recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et des conclusions de l'Inspection générale des affaires sociales exposées dans le rapport relatif à la prise en charge à l'hôpital des femmes victimes de violences. Le dispositif de cet amendement crée le cadre juridique et une incitation propice à ce que les centres d'accueil médicalisés des femmes victimes de violences soient déployés de manière concordante avec les besoins des territoires et des populations grâce à une montée en puissance des dons des particuliers et des entreprises.

des impôts. Les organismes bénéficiaires doivent présenter un intérêt général, ce qui implique qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au sens du I de l'article 206 du code précité, qu'ils fassent l'objet d'une gestion désintéressée

visant à développer, avec le concours d'associations agréées d'intermédiation locative volontaires, l'intervention des organismes d'HLM dans le parc privé. Sur le modèle du dispositif Solibail, cette proposition consiste à faire assumer des logements privés dans le diffus sur une période de dix ans par des organismes d'HLM en vue de les louer à des associations agréées d'intermédiation locative, afin de libérer des places d'hébergement dans le cadre de parcours d'insertion. Selon les chiffres du ministère du logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l'hôtel. Conformément au protocole d'accompagnement signé avec l'État en avril dernier, la contribution du mouvement HLM à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021. Cela n'est pas négligeable. Pour soutenir ce dispositif, il est proposé de soumettre les acquisitions de logements réalisées dans ce cadre par les organismes d'HLM à un droit fixe de 125 euros. L'application de ce tarif serait subordonnée

bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. Ce régime est réservé aux logements neufs. Or le mécanisme de location-accession peut également être intéressant pour les opérations d'accession sociale à la propriété

qu'il s'agit d'une démarche totalement volontaire de la collectivité, dans le cadre d'une liberté totale d'administration, nous n'avons pas de raison d'opposer un refus de principe. C'est un avis de sagesse.

Au regard de cet objectif, le monde HLM est un opérateur déterminant, parfois même le seul en territoire détendu, compte tenu de son objet social et des relations avec les collectivités locales. Le prêt d'accession sociale permet de financer environ 70 000 opérations d'accession, dont 65 % réalisés dans l'ancien et 60 % en zone rurale. Ces chiffres confirment qu'il s'agit d'un bon outil pour intervenir dans les centres-bourgs. Nous proposons donc de permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d'exonérer de droits d'enregistrement des ventes de logements qui sont réalisées dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété en centre-bourg. adopté, de conforter l'attractivité des villes moyennes en donnant la priorité à la requalification des centres anciens dégradés et en faisant revenir les habitants en centre-ville. Quel est l'avis de la commission ?

En cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d'une convention ANRU, l'article 1384 G du code général des impôts prévoit que la nouvelle construction ne peut pas bénéficier du régime d'exonération de taxe foncière prévu pour ces opérations si la construction démolie en avait bénéficié et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux. Pour favoriser les reconstructions, nous proposons que les élus locaux puissent déroger à la règle, s'ils le souhaitent.

je défends l'amendement déposé par mon collègue Antoine Lefèvre qui vise à ce que les professionnels de santé exerçant en libéral puissent bénéficier, sur décision des collectivités qui le souhaitent, d'un abattement sur la taxe foncière, comme c'est déjà le cas pour les commerces dont la superficie est inférieure à 400 mètres carrés. Un élargissement de l'abattement créé à l'occasion du projet de loi de finances pour 2018 participerait à l'effort de revitalisation des centres-villes en incitant plus de médecins à s'installer dans certaines zones, notamment dans les villes moyennes des milieux ruraux et périurbains. J'ai bien entendu ce qu'a dit le rapporteur

pour contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et lutter contre la désertification, et la majoration de taxe d'habitation pour les résidences secondaires en zones tendues, en particulier dans les grandes villes.

Ce dispositif permettrait d'avoir un outil unique, durable, plus efficace pour mobiliser les logements, alors que la crise du logement est une réalité à laquelle tous nos territoires sont confrontés, sous des formes différentes. Un outil unique permettrait de remettre sur le marché locatif des logements sous-occupés, en harmonisant le montant des impositions dues au titre des logements vacants et au titre des logements occupés en résidence secondaire, et donc de mettre fin aux effets d'aubaine entre occupation en résidence secondaire et situation de vacance, notamment dans les zones tendues. Aujourd'hui, il est plus profitable de laisser un logement vacant

plus élevé si elles le souhaitent et de préserver les mécanismes incitatifs pour la mobilisation des logements, malgré la suppression de la taxe d'habitation.

nous avons d'ores et déjà annoncé, parmi les orientations qui seront suivies, la volonté de maintenir des dispositifs à la main des élus locaux, à la fois pour sanctionner, s'ils le souhaitent, les propriétaires de logements maintenus volontairement vacants ou les propriétaires de logements qui font l'objet d'une utilisation uniquement à titre commercial, ce qui peut être

Il en est de même pour les EHPAD de statut privé lucratif qui acquittent toutefois la cotisation foncière des entreprises. Les EHPAD privés non lucratifs sont les seules composantes de l'offre d'hébergement en EHPAD

ce qui représente une rupture d'égalité devant les charges publiques pour ces structures, qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d'habilitation à l'aide sociale, et les mêmes modalités de financement. De ce fait, le moyen le plus simple pour assurer des contreparties aux retraités vivant dans les établissements privés non lucratifs serait de soumettre ceux-ci au même régime que les établissements précités en matière de taxe d'habitation. le reste à charge des résidents des établissements privés non lucratifs, qui n'acquittent pas de taxe d'habitation, augmenterait singulièrement, et un ressaut tarifaire existerait dans les EHPAD privés non lucratifs assujettis, au détriment

Une redevance est perçue par les communes concernées. Cette redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectivement de 35 %, 10 % et 55 %. La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties. La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées intéressées de la partie du tonnage extraite de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. La dernière fraction, celle de 55 %, forme, pour l'ensemble de la France, un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, du nombre de ces ouvriers ou employés. Nous considérons qu'il est nécessaire de modifier le seuil de répartition de cette troisième fraction de la redevance communale des mines. À une époque où ils étaient très nombreux, ces ouvriers et employés représentaient alors une charge pour les communes, qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l'accueil de cette population supplémentaire. Aujourd'hui, les ouvriers des mines sont moins nombreux et plus mobiles qu'avant, si bien que très peu de communes atteignent le seuil actuel de dix ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction de la redevance communale des mines, fraction la plus importante. En attendant la réforme du code minier, qui est une véritable Arlésienne depuis bien des années, nous souhaitons une répartition plus équitable du produit de la troisième fraction entre les communes minières et proposons d'abaisser le seuil pour que le premier employé ou ouvrier occupé à l'exploitation des mines et aux industries annexes déclenche cette perception.

proposons la suppression de cette troisième part, et que les crédits supplémentaires soient affectés aux deux premières tranches. En effet, les communes qui accueillent les activités industrielles minières et celles dont le sous-sol est sont les premières touchées par l'activité minière et supportent de nombreuses nuisances, notamment en termes de dégâts miniers, de risques miniers, et de développement urbain, qui perdurent bien au-delà de la période d'exploitation minière. Aujourd'hui, ces nuisances sont insuffisamment prises en compte dans la répartition de la redevance communale

passant de 55 % à 20 %, et qu'ainsi les deux autres fractions soient augmentées au bénéfice des communes dans le sous-sol est exploité, et qui connaissent de graves désordres. Quel est l'avis de la commission ?

a pour objet de tenir compte du coût des équipements collectifs permettant à ces employés de résider près de leur lieu de travail, donc les mines. Si le seuil d'attribution fixé à dix ne paraît pas, dans un premier temps, excessif, car il permet d'affecter le produit de la taxe aux collectivités ayant un nombre minimal d'ouvriers, nous sommes favorables à toute mesure qui assure une répartition plus fine entre les communes, et ce dans un objectif de péréquation. sénateur, devrait apporter un concours financier relativement limité compte tenu des critères et modes de répartition pour ces communes, dès lors que la répartition de la redevance s'effectue au prorata du nombre d'ouvriers. Nous considérons que votre proposition d'ouvrir le dispositif à des communes ayant entre trois et

mesure ne change rien pour les redevables qui bénéficient d'un dispositif d'allégement lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros. En revanche, elle évite que les collectivités territoriales ne participent à cet allégement. effet, quand il y a exonération, le prélèvement sur recettes de l'État pèse dans l'enveloppe globale des concours financiers de l'État pris en compte. Notre proposition permettrait

dispose qu'en cas de retrait d'agrément, c'est le ministre chargé de l'économie et des finances qui est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus. Cette rédaction date d'une époque où la direction générale des impôts relevait dudit ministre de l'économie et des finances. Avec cette rédaction, la DGFiP qui délivre et, le cas échéant, retire des agréments fiscaux ne pourrait pas moduler les effets de la déchéance d'un avantage fiscal qu'elle aurait elle-même accordé. Nous proposons simplement d'harmoniser la rédaction des articles 1649 et 1649 A

Cet amendement vise à créer une contribution environnementale sur les mégots de cigarettes à la charge des fabricants de tabac d'un montant de 0,2 centime d'euro par cigarette, soit 4 centimes d'euros par paquet de vingt cigarettes. vingt cigarettes. Un mégot contient 4 000 substances chimiques et met douze ans à disparaître. Il peut polluer 500 litres d'eau ou un mètre cube de neige. Près de 65 milliards de cigarettes sont fumées chaque année en France, 6 000 milliards le sont dans le monde. On ne peut plus désormais parler de lutte pour un meilleur environnement sans exiger des États qu'ils prennent des mesures draconiennes contre les mégots de cigarettes Au total, cette contribution environnementale à la seule charge des cigarettiers rapporterait 100 millions d'euros par an, une somme dérisoire par rapport au milliard d'euros de bénéfice que les cigarettiers font en France chaque année, dans le cadre de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire sans payer ni impôt ni taxe, et alors que le coût social du tabac à la charge des fumeurs et des non-fumeurs est estimé à 120 milliards d'euros chaque année ! Ces 100 millions d'euros pourraient être reversés aux collectivités locales au travers de la dotation globale de fonctionnement,

pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et pour les parcs de stationnement couverts faisant aussi l'objet d'une exploitation commerciale. Les raisons sont multiples. Premièrement, l'abattement de 50 % de la taxe d'aménagement représente une perte de recettes pour les collectivités. Dans un contexte de maîtrise des dépenses et de contraintes budgétaires, la suppression de l'abattement constituerait un apport financier important pour nos territoires. Deuxièmement, cet amendement va dans le sens de l'un des objectifs du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, adopté en 2010. La France s'est engagée à réduire progressivement, réformer ou éliminer les subventions néfastes pour la diversité biologique. Nous sommes à moins de deux ans de la fin de nos engagements, et le travail accompli est loin du résultat escompté ! Troisièmement, l'abattement de la taxe d'aménagement contribue à la consommation des sols et dessert l'atteinte des objectifs nationaux de lutte contre l'artificialisation des sols. Nous proposons en outre la publication d'un rapport par le Gouvernement visant à établir un état des lieux de l'application actuelle de la modulation de la taxe d'aménagement. Les taux de la taxe peuvent en effet être différenciés : le taux de la part communale, par exemple, se situe entre 1 % et 5 % mais peut être porté jusqu'à 20 % dans certains secteurs. Il peut également varier selon les secteurs de la commune.

? Si cet amendement était adopté, les collectivités pourraient exonérer du paiement de la taxe d'aménagement les changements de destination des locaux de production et de stockage agricoles.

de faire basculer ces dépenses de dépenses de fonctionnement en dépenses d'investissement, d'autant plus qu'elles figurent dans les comptes des régions ou des métropoles en section d'investissement.

du Gouvernement ? Nous craignons que cet amendement ne soit de nature à complexifier l'affectation actuelle de la dotation de compensation des charges transférées en section de fonctionnement, en prévoyant un dédoublement comptable et une obligation de partition de cette dotation effectuée par la commission locale d'évaluation des ressources et des charges transférées. Par ailleurs, une dotation libre d'emploi, comme le dispositif actuel, préserve la libre administration au service de transferts de compétences non conflictuels. En outre, l'adoption de cet amendement introduirait un traitement hétérogène et des inégalités de traitement, d'une part, du fait de la dégradation de la situation de l'épargne brute des métropoles qu'elle impliquerait et, d'autre part, en l'absence de dispositions similaires lors des transferts entre régions et métropoles. Enfin, cette mesure serait de nature à fausser la comparabilité des trajectoires d'évolution des dépenses de fonctionnement des départements et des recettes de fonctionnement des métropoles. Au-delà des questions de justice fiscale ou d'orthodoxie budgétaire, la disposition proposée serait un élément de complexité et serait par ailleurs assez orthogonale avec le principe même de libre administration propre à l'inscription au fonctionnement. Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable

Cet amendement a simplement pour objet de mieux cibler les contrôles portant sur le crédit d'impôt cinéma et audiovisuel de l'article 220 du code général des impôts, pour faire en sorte que le CNC ne transmette à l'administration les rapports d'audit que lorsque le rapport a identifié une irrégularité.

en relevant le tarif plafond applicable aux hôtels trois, quatre et cinq étoiles et aux palaces, et en ouvrant la possibilité pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe pour le compte

Il s'agit d'un amendement de clarification qui vise à préciser expressément dans la loi que la délibération

puisqu'à compter du 1 janvier prochain un nouveau régime de taxe de séjour sera appliqué pour les hébergements non classés. Pour être applicable, le nouveau régime impose une délibération de chaque commune et de chaque EPCI avant le 1 octobre 2018, et bien que ce ne soit pas la finalité de l'amendement, nous craignons que son adoption ne puisse conduire certaines communes et certains EPCI à se croire autorisés

C'est une demande de retrait pour les mêmes raisons. L'intention est louable- permettre aux communes de dégager un peu de trésorerie -, mais le système serait d'une complexité telle en termes de traitement et de gestion de ces versements et reversements que nous ne pouvons être favorables à ces amendements.

sur un fichier national. Ce fichier n'existera qu'à partir du mois de décembre. Dès lors, techniquement, il est impossible pour les plateformes d'adapter leur logiciel de recouvrement de cette taxe. taxe. Si l'administration, notamment celle de l'État, n'arrive pas dans les délais à fournir aux professionnels les taux et surtout aux informaticiens la possibilité de mettre leur logiciel à jour, il est difficile d'appliquer la taxe. C'est pourquoi je demande un report

à un prix de 8 euros, qui reste inférieur, par exemple, au tarif de 10 euros par nuitée à Amsterdam. Une telle disposition ne créerait donc pas une exception parisienne par rapport à d'autres grandes villes touristiques européennes, mais permettrait d'avoir un outil plus efficace.

touristiques offrent un niveau de prestations élevé, assez comparable à des hôtels haut de gamme, voire davantage. Faut-il pour autant supprimer le plafond légal de 2,30 euros ? Demeurerait alors seul le tarif le plus élevé.

est assez étonnant de vouloir modifier un dispositif avant qu'il ne soit entré en vigueur, alors que les montants, même avec le plafonnement, ne nous paraissent pas trop élevés. En ce qui concerne les deux amendements suivants, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017 a fait l'objet d'un consensus.

pour les collectivités et l'État. Il faut aussi prendre en compte le fait que l'activité hôtelière ne prive pas les habitants des villes- je pense en particulier aux Parisiens, mais c'est vrai dans l'ensemble de la métropole, comme le disait Christine Lavarde -de l'accès au logement dont chacun

s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire. À compter du 1 janvier 2019 s'appliquera une taxe de séjour proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements en attente de classement ou non classés, avons évoqué le sujet précédemment. Nous proposons d'intégrer les gîtes d'étapes et de séjour, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes au classement actuel, les soumettant au tarif applicable pour les hôtels de tourisme une étoile et assimilés,

pour les gîtes et établissements non classés, à un système fixe, comme c'était le cas antérieurement et comme c'est le cas pour les autres types de logements.

À l'échelon local, les communes du littoral agissent pour réduire l'exposition de leurs habitants à la pollution de l'air provoquée par l'industrie des ferries et des navires de croisière. Des collectivités ont développé des projets pour installer des systèmes d'alimentation électrique à quai, mais souhaitent aussi installer ce qu'on appelle des mobiles, c'est-à-dire des hottes aspirantes pour filtrer l'air contenant des particules très fines. Elles ont besoin de ressources. Aujourd'hui, le tarif applicable aux croisiéristes est celui des campings une étoile, c'est-à-dire quinze fois moins qu'un hôtel cinq étoiles. Cette nomenclature paraît en décalage avec la prestation hôtelière des navires, qui peut parfois être équivalente à celle des hôtels de haut standing. Ce problème a été soulevé en 2016 par notre collègue Gilbert Bouchet. s'agit donc de laisser un nouveau levier d'action aux collectivités, à savoir la fixation d'une taxe de séjour pour les navires les plus polluants, afin que les croisiéristes, qui viennent du monde entier, contribuent à la lutte contre la pollution de l'air. L'amendement

Dès lors qu'il s'agit d'une taxe optionnelle, il convient de rendre identifiable l'établissement assujetti à cette taxe par une mesure de publicité assurée par l'arrêté. Cela complétera le dispositif actuel par une identification des établissements et de leur répartition sur le territoire de la commune.

la collecte de la taxe de séjour ne nécessite pas d'arrêté préalable. Peut-être Michel Magras a-t-il des raisons pour demander le rétablissement des arrêtés du maire répartissant les hébergements par catégorie.

de ce projet et lui demandais s'il y aurait des problèmes de financement, celui-ci m'avait répondu : « Il y aura peut-être des problèmes de financement, car le montage financier est tout de même lié au remboursement d'une avance faite à l'industrie automobile en 2014.

rassurer. » Pour ce faire, il m'a indiqué : « Pour ce qui concerne le financement, monsieur le sénateur, c'est le Parlement, et donc vous-même, qui en a la maîtrise. Pour ma part, je fais confiance tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale pour veiller à éviter tout dérapage.

aujourd'hui 40 milliards d'euros. Bientôt, il atteindra les 60 milliards d'euros qu'avaient prévus un certain nombre de spécialistes devant la commission spéciale. Il n'y a qu'une seule source de financement,

que son coût est multiplié par deux, on va demander à des entreprises du secteur concurrentiel de mettre la main à la poche pour combler l'inefficacité des architectes de ce projet. On n'a pas d'autre solution pour ce financement.

mais il n'a pas mis le capital initial de 4 milliards d'euros. Ce soir, dans la douceur de la nuit, parce que tout va bien, que la saison va être bonne, que Noël va être bon pour les commerçants d'Île-de-France, nous allons créer deux taxes

Comme disait Pierre Dac, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites ! Ah ! Là, on dépasse les bornes. Il ne faut pas que l'Île-de-France serve de variable d'ajustement au Gouvernement pour le financement de travaux qui lui incombent. Tous les efforts ont déjà été réalisés : on fait des mutualisations dans tous les sens, on demande déjà beaucoup aux collectivités et aux entreprises dans la région. Maintenant, on crée une taxe additionnelle.

de la taille de l'agglomération parisienne et qu'ils sont satisfaisants. J'ai emprunté pendant des années le RER A, puis le RER B, tous les jours : on transporte les Parisiens

de procédure- les amendements et les suppressions d'articles -, les interrogations sur le mode de financement, sur l'affectation de la fiscalité à la métropole, aux établissements publics territoriaux, ainsi que les discussions qui les accompagnaient systématiquement sur le financement de la Société du Grand Paris. Le dispositif qui a été adopté par l'Assemblée nationale, la création d'une surtaxe égale à 15 % de la taxe de séjour, nous paraît relativement opportun dans la mesure où il permet de faire participer financièrement

alors une situation d'engorgement total de la région. Le projet est donc indispensable. Nous ne pouvons pas supprimer des possibilités de financement et ne pas résoudre ce problème. Par ailleurs, j'entends dire

que le projet est à nouveau décalé dans le temps, voire qu'il faut renoncer à des portions du projet mené par la Société du Grand Paris. Ce n'est pas très simple, mais telles sont les

des segments tout à fait particuliers de l'activité économique, dont les équilibres ne seront pas mis en cause par cette contribution supplémentaire et qui, en outre, bénéficieront, et de façon extrêmement active, de la croissance

Bon, écoutez, on n'a pas d'argent, débrouillez-vous, il va falloir faire des choix sur la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17, la ligne 18. » C'est comme cela que cela va finir. Et ce sont les collectivités territoriales qui vont devoir arbitrer entre elles. On va arbitrer entre nous

Cette taxe n'est pas satisfaisante, nous en sommes d'accord, puisqu'elle va pénaliser le secteur touristique. Augmenter la taxe de séjour dans les établissements hôteliers, c'est envoyer un très mauvais signal à un secteur économique qui exprime de vives inquiétudes. Nous venons d'en discuter. Par ailleurs, cette mesure présente un risque de contagion à d'autres régions, pourraient s'en inspirer pour financer des infrastructures. C'est pourquoi cet amendement de repli vise à limiter à deux ans la période d'application de cette taxe, à compter du 1 janvier 2019, afin de laisser à la Société du Grand Paris le temps nécessaire pour rétablir l'équilibre de ses finances

dont les bases ne sont connues qu'en mars de l'année d'imposition et les taux votés au mois d'avril de cette même année. Par conséquent, cet amendement prévoit que le produit de la taxe GEMAPI puisse être délibéré

le 15 avril. Pour cette année en particulier, qui est un peu une année charnière, il permettrait une recette aux quelques retardataires qui se sont laissés dépasser par le calendrier

Or pour notifier les bases d'imposition aux collectivités, nos services ont besoin de connaître les délibérations relatives aux institutions d'abattement ou d'exonération de taxe, qui doivent être prises avant le 1 octobre. Par conséquent, nous sommes favorables au fait d'harmoniser au 15 avril la date limite

et que les collectivités ayant mis en place la taxe spécifique pour financer cette compétence ne découvrent pas la nécessité de créer cette taxe avec l'exercice 2019, puisque cet exercice de compétence date déjà d'un an. le nombre d'intercommunalités qui seraient amenées, pour 2019, à vouloir créer la taxe et à regretter de ne pouvoir le faire avant le 15 avril me paraît limité.

Monsieur le secrétaire d'État, comment votre administration va-t-elle s'y prendre pour récupérer, au profit des collectivités qui l'auront votée, la taxe GEMAPI dans sa part taxe d'habitation qui doit disparaître progressivement dans les deux ans qui viennent ?

Les territoires d'accueil des installations du laboratoire souterrain dédié à cette recherche de gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue, il faut le dire, bénéficient d'un dispositif d'accompagnement économique spécifique, conformément à l'article L. 542-11

une taxe additionnelle aux installations nucléaires de base, dite « d'accompagnement », instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000, a été mise en place en 2007.

à écrire dans le projet de loi que les intercommunalités concernées par le périmètre des dix kilomètres pourraient percevoir également une taxe au prorata de leur population, mais définie également en décret en Conseil d'État.

en compte les problèmes d'attractivité. Si l'on considère que l'on peut taxer tous les bureaux, tous les parkings, et même tout ce qui bouge, parce qu'il faut trouver de l'argent, allons-y gaiement ! Mais, je le répète, que l'on ne vienne pas nous dire qu'il faut envoyer des missions

Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 274 amendements au cours de la journée ; il en reste 175 sur la seconde